Elle impacte également lourdement notre économie ; ses conséquences sont nombreuses : désertification du centre de la Corse, délabrement des territoires ruraux et frein à leur décisions

durée de trente ans. à l'abaissement des règles de majorité dans la gestion de l'indivision, afin que soient favorisés les règlements successoraux une fois les actes créés.

mais d'y travailler sérieusement avec la mise en place d'un groupe de travail dédié au problème du stock, qui aurait dû rendre ses conclusions au printemps, à l'aune de l'étude d'impact délivrée par le Gouvernement en mars 2017. oeuvre de ce groupe de travail.